La composition de la commission départementale de la coopération intercommunale a été modifiée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. La représentation des communes est passée de 60 % à 40 % et celle des intercommunalités de 20 % à 45 %, 40 % pour les EPCI à fiscalité propre et 5 % pour les syndicats. D'un schéma départemental de coopération intercommunale fondé par les communes, nous sommes passés à un schéma proposé par l'autorité préfectorale et modifié par les communes au sein d'une commission où leurs voix, en L'article 11 de cette proposition de loi supprime certes le pouvoir de modification de ces schémas par les CDCI ; il est néanmoins proposé de revoir la composition de la CDCI, afin d'y assurer une plus grande représentation des maires et des élus municipaux. Naturellement, madame la ministre, vous le comprenez, mon amendement

mais qu'il n'était pas question de revenir sur le mode de scrutin dans les intercommunalités, ou EPCI, classiques. Nous voici rassurés !

L'article 11 de la proposition de loi modifie en profondeur les pouvoirs de la commission départementale de la coopération intercommunale. Afin de conforter le rôle des communes, qui constituent la cellule de base de la démocratie locale, dans le fonctionnement de l'intercommunalité, nous proposons de prévoir que la CDCI se réunit au moins une fois par an.

de vote. Je comprends parfaitement que l'on n'oblige pas les EPCI à créer des réunions des maires.

d'une commune qui aurait pour conseil municipal la somme des conseils municipaux ! On essaye de se battre pour que les intercommunalités fassent leur boulot d'intercommunalité et que les communes puissent continuer à faire leur

L'objectif est tout simplement de faire en sorte que le parlementaire soit beaucoup plus proche des décisions tout à fait structurantes de son territoire et ait voix consultative au sein de la CDCI.

une question très importante. Nous nous sommes prononcés cet après-midi sur une autre proposition de loi visant à permettre à tous les parlementaires du département d'assister à la commission départementale de la coopération intercommunale.

à ne pas avoir le droit de rendre ce genre de services à la collectivité. Pour autant, j'ai la faiblesse de penser que, en raison de notre expérience, nous ne sommes pas forcément les moins qualifiés.

reconnue par la loi, les parlementaires doivent tout de même s'efforcer de rester présents au coeur de leur département, et de défendre les communes et les intercommunalités pour la

d'étude d'impact. En l'occurrence, il s'agit de l'obligation pour les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants de s'inscrire en préfecture.

Nous avions alors constaté que, dans certaines communes, en particulier dans mon département, des candidats aux élections municipales se trouvaient sur des listes sans qu'ils aient donné leur approbation pour y figurer. avions donc introduit, en plus de la déclaration de candidature, la nécessité d'authentifier celle-ci par la fourniture d'une photocopie de pièce d'identité et l'apposition d'une signature.

un argument de bon sens : la garantie pour l'électeur que le candidat est bien candidat et qu'il n'y a pas de supercherie. Enfin, pour ce qui concerne les conseils municipaux incomplets, nous avions introduit à l'époque par le

Comme Pierre-Yves Collombat, je pense que, lorsqu'on souhaite être élu, il faut se porter candidat et le formaliser, de la manière la plus simple, en faisant vérifier son identité par l'autorité locale la plus adaptée, c'est-à-dire la préfecture.

de confier au citoyen électeur le soin de déterminer lequel de ses voisins était le plus à même d'exercer une responsabilité.

de nombreux maires lui raconter toutes les difficultés qu'ils éprouvent à constituer des listes. Ils vont à la pêche aux candidats et réussissent à boucher les trous grâce à la bonne volonté de

Les principaux objectifs de la réforme de 2013 étaient de renforcer la parité, ce qui est louable, d'améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités et de les rendre plus lisibles pour les citoyens. Si le premier objectif a naturellement été atteint, les deux autres ne le sont pas. En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et complexifie parfois même la gestion municipale. Les aléas de la vie municipale font qu'un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte : les conseillers communautaires sont le maire, les adjoints, puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. Or cette exigence n'a pas de réelle justification. Ah si ! En effet, il n'existe aucun lien entre la composition d'un exécutif municipal et les compétences de l'intercommunalité. Ainsi, pendant les mes trois premiers adjoints successifs étaient délégués à l'action sociale- quand on est gaulliste, on ne se refait pas ... Selon quels principes un maire devrait-il définir l'ordre de ses adjoints et leurs délégations en fonction de l'intercommunalité ?

pour financer les bureaux d'études. Il apparaît donc nécessaire que les départements, garants de la solidarité territoriale, étendent ou diversifient leurs services d'ingénierie auprès des communes et des EPCI de moins de 50 000 habitants, dans le but de renforcer le développement des politiques et projets locaux.

au Conseil d'État. Il a pour objet d'adapter le champ des compétences couvertes par l'assistance technique des départements, afin de tenir compte des extensions décidées par le législateur. Par ailleurs, le

de notre collègue, mais aussi de régler tous les problèmes de concurrence déloyale qui pourraient être soulevés.

est satisfait, puisque l'État peut déjà déléguer toute compétence qui lui est propre à une collectivité territoriale et qu'en l'espèce,

Il n'en existe que deux en France, en Isère et dans le Nord, mais légalement, les conseillers de ces deux EPCI sont actuellement privés d'indemnités. J'avais une pensée pour eux, et je ne suis pas le seul Plus généralement, je proposais de revaloriser les indemnités des maires et des adjoints des communes les plus petites, par une meilleure progressivité. Après l'adoption, dans la loi de finances pour 2018, d'un article augmentant l'indemnité des maires des grandes villes de 40 %, cela ne me paraissait tout de même pas extravagant d'envisager un parallélisme des formes. Les maires ne comprendraient pas que nous n'allions pas plus loin que la modeste revalorisation de l'indice. Véritables bénévoles de la République, près de 20 000 maires des communes de moins de 500 habitants ne perçoivent que 658 euros bruts par mois, malgré l'augmentation de leurs responsabilités ... et- il faut y penser Enfin, dans les EPCI, tous les maires ne peuvent pas occuper la fonction de vice-président. En découle une différence d'indemnisation importante entre les maires, qui peuvent parfois subir un chantage au maintien de leur délégation et, donc, de leurs indemnités. Il convient ainsi de réfléchir à renforcer l'indépendance des maires.

de séances de questions orales réservées à l'opposition, afin que celle-ci puisse exercer un contrôle sur les actes de la majorité. Il est proposé de réécrire cet article afin de fixer une règle générale pour ce droit aux questions orales.

invite un certain nombre de présidents d'exécutif à revenir sur ces accords trouvés entre tous les groupes politiques de la collectivité et à en rabattre sur les droits, principalement de l'opposition.

Belenet. Toutefois, et c'est un constat partagé, les indemnités des maires et adjoints des petites communes étant relativement faibles, la commission a jugé préférable de ne pas les soumettre à ce prélèvement. Elle émet donc un avis défavorable.

traduit la volonté de mettre en place un système mutualiste bénéficiant à tous les élus locaux, mais dont le financement est assuré par eux-mêmes, sur leurs indemnités de fonction, et non tiré des budgets des collectivités territoriales.

Sur le modèle des dispositions existantes pour les départements et les régions introduites par l'article 107 de la loi NOTRe, je propose d'étendre aux EPCI de plus de 10 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, l'obligation d'annexer à leur compte administratif un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice. Comme la commission l'a adopté, à l'article 20 de la proposition de loi, pour les départements et les régions, cet état récapitulatif sera ensuite mis en ligne sur le site internet de l'EPCI. Il s'agit là d'une mesure de transparence de l'action communautaire.

madame la ministre

le principe même d'un statut de l'élu. Il reviendra aux travaux en cours de l'alimenter, de le compléter,

Cet amendement vise à supprimer une bizarrerie

les indemnités de fonction sont attribuées de manière forfaitaire, sans relation avec le temps que l'élu consacre à l'exercice de ses fonctions. Un élu local n'est pas assujetti à un contrat de travail. Il exerce une mission pour laquelle il s'est porté candidat. Ainsi,

Madame la ministre, si les raisons que vous avancez sont si importantes que vous voulez bien le dire, je ne vois pas pourquoi une réflexion plus approfondie les ferait disparaître

est tout de même important d'avoir la notion des proportions ... Pour cette armée de soldats de la République que sont les élus locaux, je suis très fier et très heureux que l'on conserve